Monsieur le président, madame la rapporteure générale- chère Élisabeth Doineau

Pour autant, je ne peux évidemment que regretter le fait que vous n'adoptiez pas ce texte qui, je le crois sincèrement, permet de soutenir notre système de santé, d'ouvrir plus de droits à nos concitoyens, et acte une réforme profonde du champ de l'autonomie. Avec ce texte, nous parachevons en effet une étape essentielle de la réforme du soutien à l'autonomie, en transformant radicalement l'offre à destination des personnes en perte d'autonomie et en amorçant la création du service public de l'autonomie tel qu'il a été évoqué par le Président de la République dans sa dernière allocution. d'une réforme ambitieuse, qui repose sur 1,3 milliard d'euros de mesures nouvelles d'ici à 2025 et qui est financée par les moyens d'ores et déjà rendus disponibles pour la branche autonomie à l'horizon de 2024. Cette réforme structurelle se fera avec les départements, que nous accompagnerons au cours de ces transformations. Nous investissons d'abord pour renforcer la lisibilité et la qualité de l'offre de services à domicile et nous garantissons une plus grande équité dans le financement des structures selon les territoires, d'un tarif national de référence pour la tarification des interventions à domicile, d'une dotation complémentaire au service de la qualité des services à domicile

d'un grand chantier de simplification et de fusion de services visant à créer le « service autonomie à domicile », interlocuteur unique des personnes âgées en perte d'autonomie. Assumer ce choix en faveur du domicile nous permet, par la même occasion, de porter une réforme transformatrice pour nos établissements, afin d'adapter ces derniers à l'accueil de personnes d'un âge de plus en plus avancé.

et nous engageons le remboursement des consultations d'un psychologue. Nous consacrons ces droits nouveaux par la solidarité nationale, tout en tirant les leçons de la crise sanitaire. Ainsi, nous accélérons l'innovation en santé, nous renforçons notre souveraineté pharmaceutique et- je crois que nous pouvons tous nous en féliciter -nous favorisons l'accès aux droits sociaux des Français.

d'éviter toute iniquité entre deux soignants exerçant le même métier mais dans des structures financées par des acteurs différents. Cette philosophie s'appliquera également aux résidences autonomie, dont tous les soignants verront leur rémunération revalorisée grâce au Ségur

deux avancées importantes, pour lesquelles de nombreux parlementaires s'étaient mobilisés : l'extension à 24 ans de l'âge jusqu'auquel les enfants majeurs peuvent bénéficier du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle comme ayant droit de leurs parents, ce qui permettra de garantir un meilleur accès des jeunes aux soins ; et la mise en place d'un capital-décès pour les familles des non-salariés agricoles, qui permettra d'apporter un soutien financier à ces familles lorsqu'elles sont confrontées au décès d'un des leurs d'une maladie, d'un accident de la vie privée ou d'un suicide. Ce sont de belles avancées, que votre travail et votre mobilisation auront permis d'intégrer dans ce texte pour améliorer l'accès aux soins et la protection de nos concitoyens. La parole

; la suppression du plafonnement de la participation de la CNSA au financement des dépenses induites, pour les départements, par l'avenant 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile, adoptée sur l'initiative du rapporteur pour la branche autonomie, Philippe Mouiller

ou encore l'extension du droit à un capital-décès aux ayants droit des non-salariés agricoles, adoptée sur l'initiative conjointe de Françoise Férat, d'Henri Cabanel et du Gouvernement. Pour autant, à mes yeux, le compte n'y est pas, loin de là, et les différences entre le texte soumis en nouvelle lecture et celui que nous avons adopté en première lecture sont considérables. Tout d'abord, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 23, qui approuve l'annexe B du PLFSS. Certes, ce rétablissement d'un article obligatoire d'une loi de financement est logique, ne serait-ce que pour assurer la régularité du texte, mais il est décevant, dans la mesure où cette annexe ne prévoit toujours pas de stratégie de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale après la crise. De plus, même en tenant compte de l'amélioration de la conjoncture économique, la trajectoire financière de l'annexe B fait toujours apparaître un plateau de déficit à un niveau insoutenable à l'horizon de 2025-

Cet article reste donc inacceptable, même dans sa nouvelle rédaction. Pourquoi l'équilibre représente-t-il un objectif impérieux ? Parce que, par définition, le déséquilibre est inconfortable sur la durée. La dette corsète, anéantit, obère, réduit toute forme de générosité à l'avenir.

et, d'autre part, que l'on ne peut pas mélanger n'importe quoi avec la dette sociale si l'on ambitionne vraiment d'apurer celle-ci un jour. Dans cette logique, le Sénat s'oppose encore plus au financement par la Cades d'investissements nouveaux et ne et ne pourra donc accepter le retour de l'article 5. La Caisse n'est pas un fonds d'investissement ! Par ailleurs, l'Assemblée nationale a supprimé les mesures adoptées par le Sénat afin d'améliorer l'équilibre de l'année 2021. Il en est ainsi de l'augmentation du rendement de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM). Il en va de même de l'amendement tendant à prévoir la compensation intégrale, pour la sécurité sociale, du coût de la subvention (Santé publique France), qui a explosé pour la deuxième année consécutive, toujours sans la moindre consultation du Parlement. De manière plus structurelle, l'Assemblée nationale a également supprimé l'article 58 que le Sénat avait introduit sur l'initiative du rapporteur pour la branche vieillesse, René-Paul Savary. Je le rappelle, cet article prévoyait la convocation d'une conférence de financement réunissant les représentants des organisations syndicales des salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l'État, pour formuler des propositions destinées à ramener à l'équilibre financier l'ensemble des régimes de retraite de base en 2030. Ce dispositif prévoyait également que, à défaut d'accord, des mesures paramétriques entreraient en vigueur au 1 janvier 2023, relatives à l'âge de départ, à la durée de cotisation et à l'alignement des régimes spéciaux. Enfin, les députés ont rétabli de nombreux articles que nous qualifions de « cavaliers sociaux », car ils sont étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale, et ont été introduits dans ce texte simplement pour masquer l'absence d'une véritable loi Grand Âge ou d'une loi sur les professions de santé. Je conclurai en faisant une observation particulière sur les amendements identiques, à l'article 54, émanant de la commission et de Jean-Marie Vanlerenberghe, ancien rapporteur général

je me permets de vous le dire, madame la ministre, il augure très mal de la possibilité d'obtenir un accord de commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. mes chers collègues, que, au moment de cet examen, nous sommes en quelque sorte parvenus au terme du dialogue utile entre les deux assemblées dans le cadre de cette navette. C'est la raison pour laquelle, au vu de la profondeur des divergences qui subsistent, la commission des affaires sociales, qui s'est réunie ce matin, proposera au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Il s'agit d'un texte important, ambitieux, puisqu'il traduit les engagements du Gouvernement pris dans le cadre du Ségur de la santé et les revalorisations salariales historiques décidées Une nouvelle fois, l'examen du PLFSS est un moment charnière pour notre pays, car ce texte consacre de nombreuses avancées répondant aux attentes des Français dans toute leur pluralité. Je pense notamment à la possibilité de se faire prescrire des lunettes chez un orthoptiste, alors que, nous le savons, le délai moyen d'attente chez les ophtalmologues atteint six mois. également à la généralisation de la télésurveillance pour les 20 millions de Français atteints de maladies chroniques, afin de renforcer la prise en charge effective de ces patients, ainsi qu'à l'octroi automatique de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et à la simplification de son attribution aux bénéficiaires du minimum vieillesse. Je pense, enfin, au remboursement à 100 % de la contraception pour les 3 millions de femmes âgées de moins de 26 ans, véritable mesure de justice sociale, puisque les études montrent que l'achat de moyens de contraception est le plus souvent le fait des femmes.

Pour autant, nous sommes conscients des désaccords qui persistent entre les deux chambres. Nous les entendons et nous les respectons, car ils constituent l'intérêt même du débat législatif. Cette nouvelle lecture aurait permis d'en débattre.

ou encore l'assouplissement des conditions de dispensation, par le pharmacien, de produits de santé aux patients atteints de maladies chroniques après expiration de l'ordonnance. Oui, l'Assemblée nationale a apporté des modifications, et c'est son rôle. Mais cela aurait pu aussi être le nôtre aujourd'hui. Nous nous félicitons ainsi de la réintroduction de l'article 5, essentiel à nos yeux. De même, la réintroduction du rapport sur la contraception masculine ou encore la suppression de la énième réforme des retraites déguisée sont des modifications que le groupe RDPI Un certain nombre de dispositions que nous promouvions ont été adoptées conformes à l'Assemblée nationale. Ainsi, nous nous félicitons que les exigences d'interopérabilité applicables aux dispositifs médicaux aient été maintenues,

ce PLFSS est d'autant plus essentiel que la cinquième vague nous rappelle l'épidémie qui persiste et l'engagement de tous face à celle-ci. Nous pensons que le budget de la sécurité sociale mérite mieux qu'une énième manoeuvre politicienne, mais nous devons nous en remettre, à contrecoeur, au travail de nos collègues députés ... Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur, une délégation conduite par M. Bodo Ramelow, ministre-président du Land de Thuringe et président du Bundesrat allemand. Elle est accompagnée par nos collègues Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères et de la défense, et Ronan Le Gleut, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Allemagne, ainsi que par son excellence M. Hans-Dieter Lucas, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en France. La délégation a été reçue ce matin en audience puis à déjeuner par le président Gérard Larcher. Cette rencontre entre les présidents du Bundesrat et du Sénat s'inscrit dans le cadre d'une coopération étroite et de longue date. Un nouvel élan a été donné à la relation entre les deux institutions par la signature, le 19 mars 2019, d'une déclaration commune entre le Sénat et le Bundesrat, dans le contexte de la nouvelle orientation donnée à la relation franco-allemande par le traité d'Aix-la-Chapelle. Cette coopération se poursuit, dans le cadre du « triangle de Weimar », avec le Sénat de Pologne. Partageant de nombreux sujets d'intérêt commun, notamment en matière de questions européennes, de coopération décentralisée et transfrontalière et de subsidiarité, le Sénat et le Bundesrat apportent une contribution essentielle à la relation entre la France et l'Allemagne. La visite du président du Bundesrat est ainsi l'occasion de manifester le profond attachement du Sénat à l'amitié franco-allemande et à son rôle majeur au sein de l'Union européenne. Les travaux conjoints entre nos deux institutions se poursuivront très prochainement, dans le cadre de la vingt et unième rencontre des groupes d'amitié du Sénat et du Bundesrat, qui se tiendra à Berlin, à l'invitation du Bundesrat, du 9 au 11 décembre prochains, et dans le cadre du volet parlementaire de la présidence française de l'Union européenne, qui débutera le 1 janvier 2022, au cours de laquelle le couple franco-allemand aura un rôle éminent à jouer. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à M. Bodo Ramelow et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat français.

la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 n'est pas parvenue à un accord. Les divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale portent essentiellement sur trois points : la question des retraites,

En dépit de ces divergences, l'examen du texte par le Sénat a permis d'apporter des améliorations bienvenues. Je suis en effet favorable au dispositif de conventionnement sélectif des médecins après six mois de remplacement dans un désert médical,

ainsi qu'un amendement visant à astreindre les jeunes médecins diplômés à exercer, pendant un an, dans un désert médical. Le développement de la télémédecine peut apporter des solutions complémentaires. Les mesures de revalorisation salariale issues du Ségur de la santé pourront bénéficier à l'ensemble du secteur médical et médico-social, ce qui représente une avancée importante. L'automatisation du versement des pensions alimentaires, destinée à limiter les risques d'impayé, et la prise en charge de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans représentent

aux personnes âgées vivant à domicile et souffrant de troubles cognitifs. Ce dispositif aurait été très facilement applicable. Malheureusement,

soignants, dans un contexte d'augmentation du degré de dépendance globale, qui se situe en moyenne à près de 750

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Gouvernement revient, en nouvelle lecture, devant la Haute Assemblée avec un projet sensiblement identique à celui qui nous a été transmis en première lecture. Même si ce n'est pas une surprise pour nous, nous regrettons que le Gouvernement et sa majorité aient balayé la quasi-totalité des propositions du Sénat. Nous avions fait le choix de prendre nos responsabilités, afin de préserver à long terme la solidité de notre modèle social. Telle a été notre boussole pour la branche vieillesse : équilibrer notre système de retraite par répartition, auquel nous sommes tous attachés. Avec un déficit qui devrait atteindre 10 milliards d'euros d'ici à 2025, il est urgent non pas d'attendre mais d'agir ! C'est la place des seniors dans notre société qui est en cause. Il est vrai que plusieurs solutions peuvent théoriquement être choisies pour ramener notre système de retraite à l'équilibre, mais nous avons toujours écarté la diminution des pensions et l'augmentation des cotisations nous estimons que le recours à la dette n'est pas une solution, car celle-ci devra tout de même être remboursée par les générations futures. La dette compromet le principe même de la répartition. Dès lors, seuls le report de l'âge de départ à la retraite et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, ainsi que le Sénat l'avait proposé, sont à même de prévenir le désastre annoncé et d'éviter la paupérisation des retraités. Cette perspective financière de la branche vieillesse est d'autant plus inquiétante que la baisse de la natalité se confirme année après année. Moins de naissances aujourd'hui, c'est moins d'actifs demain pour cotiser. Aujourd'hui, on dénombre 2,1 actifs pour un retraité ; en 2040, il n'y en aura plus que 1,5, mais, avec une baisse de la natalité plus forte que prévu, ce ratio pourrait encore s'aggraver. Il est donc regrettable que la branche famille fasse l'objet, une fois encore, de si peu de mesures dans le PLFSS, alors que la politique familiale dans notre pays a besoin d'une renaissance. Ce manque de mesures ambitieuses est incompréhensible au regard de la situation de la branche. On mesure les conséquences sur la politique familiale du fait de n'être pas revenu sur l'universalité des prestations. Le défaut de mesures est également évident lorsque nous examinons la branche autonomie. Les constats et les besoins sont connus depuis plusieurs années. Or cette branche achève son premier exercice en déficit, lequel devrait doubler en 2022 pour s'établir à 900 millions d'euros. Cette situation ne devrait connaître aucune amélioration avant l'affectation à la branche, en 2024, d'une fraction de la CSG. Nous avons approuvé l'extension des mesures du Ségur secteur médico-social, mais cette politique des petits pas visant à ajuster au coup par coup des mesures en faveur du personnel provoque des incompréhensions et ne fait qu'aggraver les difficultés de recrutement rencontrées dans de nombreuses structures. La question du financement de la perte d'autonomie ne trouve pas non plus de réponse dans ce PLFSS. Afficher une branche autonomie à crédit, c'est remettre en cause une politique de l'autonomie fondée sur une solidarité intragénérationnelle. En matière de santé, nous

Si nous comprenons l'intention du Gouvernement de faciliter l'accès direct à certains professionnels, nous considérons que ces mesures, tout en remettant en question le parcours de soins et le rôle du médecin référent, auraient plutôt trouvé leur place dans une loi Santé. Par ailleurs, en matière de déficit de l'offre médicale, l'amendement que le Sénat a adopté n'avait qu'un seul objectif : ne pas mettre en place un conventionnement sélectif, ce qui reviendrait à supprimer encore davantage la liberté d'installation. Là encore, il est urgent d'agir : la colère monte, l'exaspération s'amplifie ! L'ensemble des territoires est concerné par le manque de médecins. Le fait que plus de 8 % de la population,

au minimum un stage d'un semestre ... »- et non d'un an, mon cher docteur Chasseing -« ... en pratique ambulatoire. Ce stage [ ...] est effectué sous un régime d'autonomie supervisée ». Chaque année, plus de 3 900 internes pourraient donc exercer dans les territoires.

favoriser l'installation de médecins dans les zones sous-dotées. C'est l'une des premières préoccupations, à juste titre, de nos concitoyens et des élus. Par ailleurs, certaines mesures votées dans le cadre de ce texte doivent nous interroger sur la définition même d'une loi de financement de la sécurité sociale. Trois principes doivent prévaloir dans la répartition des actes médicaux entre médecins, spécialistes ou non, et paramédicaux, dans le respect du médecin référent.

tout acte médical ou paramédical engage la responsabilité non seulement de son effecteur, mais aussi de son prescripteur. Ce n'est donc pas à travers des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale

utiliser le système social de remboursement en fonction de ses besoins et payer en fonction de ses moyens ; pour la branche vieillesse, les cotisations des actifs actuels servent à payer les pensions des retraités d'aujourd'hui.

nationale. Avec ce PLFSS, le bicamérisme français devient un fantôme. Cette année encore, la loi sera écrite par Emmanuel Macron et aucune objection n'aura été entendue, certainement pas celles du Sénat, renvoyé au silence de façon quelque peu insupportable. Sur le fond, qu'avons-nous donc à dire d'un texte qui ne semble pas nous appartenir sinon que, encore une fois, les Ondam prévisionnels des établissements de santé sont inférieurs aux besoins réels et que les hôpitaux semblent condamnés à la crise perpétuelle. En témoignent les restructurations brutales qui privent de soignants, de lits et d'hôpitaux de proximité des territoires entiers : 25 établissements étaient fermés l'an dernier, de même que 5 700 lits d'hospitalisation complète, tandis que les soignants en première ligne continuent de se battre contre le covid. À la dette des hôpitaux se conjuguera celle, organisée,

la qualité du soin dû à toute personne en perte d'autonomie. Cela résulte finalement d'une logique que la philosophe Joan Tronto, théoricienne féministe du « care », résumait en ces termes : « Pourquoi ne respectons-nous pas les personnes qui prennent soin des gens, des animaux et de l'environnement autant, sinon plus, que les personnes qui font et gèrent l'argent ? Parce qu'il existe, dans nos sociétés, une compétition, entre la logique de la richesse capitaliste et celle du " soin ", et jusqu'à présent, en tant que société, nous nous sommes continuellement rangés du côté de la richesse. Bien sûr, nous nous réjouissons de l'extension du Ségur au secteur du médico-social et à celles et ceux qui en avaient été arbitrairement exclus. Nous saluons également les nouvelles dispositions, retoquées ici même, visant à promouvoir la prise en charge de la contraception masculine : il s'agit d'une avancée vers un partage réel de la charge mentale liée à la contraception.

Nous restons aussi conscientes et conscients du chemin immense qui reste à parcourir pour sortir les politiques de santé des rivets de l'austérité et des préoccupations avant tout économiques, et pour construire enfin une démocratie écologique du soin. Si nous actons donc certaines avancées du projet de loi, nous en récusons la forme qui semble faire fi du bicamérisme démocratique, et nous en récusons surtout la logique austéritaire qui se refuse à aller chercher les ressources nécessaires au redressement durable de l'hôpital, à la lutte contre l'intensification de la

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que la pandémie de covid-19 repart en flèche, j'ai une pensée pour l'ensemble des personnels des hôpitaux qui doivent, en sous-effectifs, et en ressentant une forme de déconsidération de la part des directions d'établissements et du Gouvernement, Malheureusement, ce budget de la sécurité sociale pour 2022 ne répond pas plus que le Ségur de la santé à l'urgence de la situation. Il ne prévoit aucune mesure pour rattraper le retard ni investir dans l'avenir.

Le déficit de 15 milliards d'euros de la sécurité sociale à l'horizon 2025 est sciemment organisé : on agite un chiffon rouge pour mieux justifier les futures économies, déjà programmées. C'est ainsi que la majorité sénatoriale a motivé le report à 64 ans de l'âge de

À l'inverse du projet gouvernemental et de celui de la majorité sénatoriale, nous portons un projet politique qui rétablit la justice sociale et qui met le capital à contribution. Ainsi, nous proposons de supprimer les 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales pour les investir dans un grand plan de renforcement du service public hospitalier, avec le recrutement de 100 000 personnels. Nous proposons également de mettre à contribution les revenus financiers afin de créer un grand service public de l'autonomie,

pour financer un pôle public du médicament et des produits de santé qui garantisse notre souveraineté sanitaire et l'arrêt des pénuries de médicaments. Parallèlement, nous défendons, à l'échelle européenne, la levée des brevets et des droits de propriété intellectuelle pour garantir l'accès de l'ensemble des peuples au vaccin contre la covid-19, bien commun de l'humanité. Je vous appelle d'autant plus à agir en ce sens, madame la ministre, qu'avec la quatrième dose de vaccination, c'est le jackpot assuré pour quelques grands Enfin, nous proposons de lutter véritablement contre la fraude patronale aux cotisations sociales et d'investir ces 80 milliards d'euros pour augmenter le nombre de professionnels formés et développer des centres de santé dans chaque département, afin de lutter contre les déserts médicaux. Ce PLFSS n'a rien d'exceptionnel, malgré vos grands grands et beaux discours. Il poursuit les mêmes logiques et prévoit les mêmes remèdes qui font que l'hôpital, le secteur médico-social et notre système de santé et de protection sociale sont aujourd'hui à bout de souffle.

sont saturés et nous connaissons de gros problèmes pour recruter des personnels médicaux et paramédicaux. Malgré tout, vous avez continué, en pleine crise, de fermer 5 700 lits. Changer totalement de logique est une urgence pour améliorer les conditions de travail des soignants, afin de les fidéliser et aussi de faire revenir celles et ceux qui ont quitté l'hôpital découragés, épuisés ... Caroline Brémaud, cheffe de service des urgences du centre hospitalier de Laval, m'a dit, à juste titre, que le premier médicament pour soulager un patient était l'humain, le temps passé aux côtés des malades plutôt qu'à remplir des tableaux ou à codifier ! C'est parce que ce PLFSS 2022 ne lui en donnera pas les moyens, ni à elle ni à aucun autre de ses collègues, que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera contre ce projet de budget de la sécurité

comme chaque année, nous voilà contraints de nous réunir à nouveau pour étudier ce projet de loi de financement de la sécurité sociale après l'échec de la commission mixte paritaire. Le sentiment du groupe Union Centriste, après ce nouvel échec des discussions avec l'Assemblée nationale, est plus que mitigé. Nous nous interrogeons notamment sur la capacité du Gouvernement à écouter une voix différente de la sienne. Nos divergences politiques sont nombreuses et nous voyons un clivage clair entre nos deux assemblées : une façon différente d'aborder le débat sur les finances de notre sécurité sociale. Nos critiques sur ce texte sont, elles nous ne nous en sommes pas cachés en première lecture. Je souhaite en relever quatre aujourd'hui. Tout d'abord, nous déplorons un projet peu ambitieux, muet sur les perspectives financières de la sécurité sociale, et, pire encore, qui ne propose aucune solution pour sortir de la dette abyssale dans laquelle est plongée notre assurance maladie. Il nous semble urgent de définir une stratégie de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale après la crise. C'est le sens du vote de suppression de l'article 23 par notre assemblée, sur la proposition de Mme la rapporteure générale : maintenir jusqu'en 2025 un déficit de plus de 10 milliards d'euros est inenvisageable. Nous avons la responsabilité d'agir sur cette question. C'est

concerne la reprise de la dette hospitalière par la branche maladie. Nous partageons le constat du Gouvernement sur la nécessité d'engager les établissements assurant le service public hospitalier dans une trajectoire vertueuse de désendettement et d'investissement. Mais ce n'est pas à la sécurité sociale d'éponger leurs dettes : c'est le Enfin, notre quatrième opposition a pour objet le transfert financier entre les branches famille et maladie- René-Paul Savary l'a rappelé -, visant à compenser la prise en charge par cette dernière des indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants.

Notre démographie est en berne. Les jeunes parents ne trouvent pas le mode de garde adéquat pour leurs enfants. Le modèle de la famille française évolue : il a besoin du soutien de l'État et d'une véritable politique ambitieuse, qui accompagne et qui donne un cap. Si le Gouvernement préfère regarder ailleurs et réorienter les financements de nos aides publiques aux familles, tel n'est pas notre choix ni celui du Sénat. Nous regrettons enfin que plusieurs amendements particulièrement intéressants, déposés par notre groupe, ne figurent pas dans la version finale du texte. Je pense notamment à l'extension des des garanties complémentaires au risque de perte d'autonomie chez un proche, portée par Jocelyne Guidez, à la pérennisation de l'exonération de cotisation spécifique à l'emploi de travailleurs saisonniers demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole, portée par Valérie Létard, et à la dérogation à la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur,

parmi lesquels la quasi-totalité des articles récapitulatifs. Nous avons conservé l'esprit de nombreux autres articles. Parmi ces points d'accord figurent l'amélioration de l'indemnisation des victimes professionnelles de pesticides, l'extension des revalorisations du Ségur de la santé aux personnels du secteur médico-social, le tarif plancher national pour les services à domicile, la revalorisation et l'extension de l'allocation journalière du proche aidant ou encore l'assouplissement du cumul emploi-retraite pour les soignants mobilisés pendant la crise sanitaire. Pour ce qui concerne la branche famille, dont j'ai la responsabilité, le Sénat a adopté la généralisation de l'intermédiation des pensions familiales. De même, dix-huit amendements du Sénat ont été repris dans le texte de l'Assemblée nationale, dont un seul avait été adopté contre l'avis du Gouvernement. Nous nous félicitons notamment que l'amendement de notre collègue Françoise Férat concernant l'extension du droit à un capital décès aux ayants droit

notamment au rejet du financement de la dette hospitalière par la Cades ou encore à la réforme paramétrique du système de retraite. Sans surprise également, l'Assemblée nationale a, cette année encore, rétabli l'essentiel du texte qu'elle avait adopté en première lecture. C'est la raison pour laquelle la commission nous proposera, dans quelques instants, d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable. la troisième fois cette semaine que notre assemblée, pourtant reconnue pour la richesse de ses échanges, refusera de débattre. Le groupe RDSE déplore profondément ce positionnement qui aboutit à un monocamérisme de fait. Ce PLFSS comporte pourtant un certain nombre de mesures positives, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un consensus entre nos deux assemblées. Je pense, par exemple, à l'extension des revalorisations du Ségur de la santé aux personnels du secteur médico-social,

pour la rémunération des personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile, à la prise en charge intégrale de l'ensemble des frais liés à la contraception pour les femmes de moins de 26 ans, même si nous regrettons que la mesure n'ait pas été étendue à la contraception masculine. l'accès direct à certains professionnels de santé. Comme l'a rappelé ma collègue Véronique Guillotin, la médecine de ville est en crise et ces expérimentations permettront de libérer du temps médical. L'expérimentation de la prise en charge de substituts nicotiniques délivrés par les pharmaciens sans ordonnance est une bonne chose, alors que le tabagisme reste la première cause de décès évitable. Je pense, la suppression de la surcotisation salariale sur la prime de feu versée aux sapeurs-pompiers professionnels. Cette disposition avait été adoptée par le Sénat dans le PLFSS pour 2021 avant d'être rejetée, à l'époque, par nos collègues députés. certaines dispositions introduites au Sénat ont été maintenues par l'Assemblée nationale. Je pense tout particulièrement à la mise en place d'un capital décès, destiné à apporter un soutien financier aux familles des non-salariés agricoles, lorsqu'elles sont confrontées au décès d'un des leurs après une maladie, un accident de la vie privée ou un suicide. Cette mesure est une avancée significative pour l'accompagnement des agriculteurs en détresse, sujet porté depuis longtemps par notre collègue Henri Cabanel.

l'extension aux EPCI du bénéfice des exonérations de cotisations patronales sur l'emploi d'aides à domicile ; l'alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes ; ou encore la mise en place d'une taxe sur la publicité en faveur des jeux d'argent en ligne ... Je pense également à la création de zones franches médicales, levier supplémentaire pour lutter contre la désertification médicale. Pour autant, nous regrettons une nouvelle fois que cette ultime discussion ne puisse avoir lieu au sein de notre assemblée. Je le répète, le RDSE est profondément attaché au débat entre les deux chambres, à chaque fois que cela est possible.

Aussi, le texte qui nous revient confirme le maintien d'une sécurité sociale structurellement déficitaire, ce que nous regrettons. Le maintien de cette dette continue de transmettre un message politique négatif, celui d'un système de protection sociale qui coûterait trop cher. En cela, la création d'une branche autonomie originellement déficitaire nous interroge sur le sens que souhaite donner le Gouvernement à cette cinquième branche.

et ce en dépit de toutes les contestations des professionnels visés à travers un corpus d'articles dont la plupart ont été ajoutés par voie d'amendement, nous constatons une fois encore un problème de méthode et de vision qui consiste à imposer, verticalement, un bouleversement de notre système de soins et des rapports entre professionnels de santé. Certes, nous avons dit que des évolutions étaient nécessaires, mais elles nécessitent une concertation en profondeur et un dialogue interprofessionnel nourri qui, seuls, permettent de contribuer à une amélioration de l'accès aux soins. Le retour à la mouture initiale du texte de l'Assemblée nationale sur presque tous ces articles témoigne d'un manque de considération pour les corps intermédiaires, contribuant à des tensions entre professionnels et ne permettant pas d'avancer collectivement dans le même sens.

Au lieu d'établir des réformes d'ordre structurel, dont la pandémie a permis de souligner le besoin, ce budget s'attache à perpétuer, sans les remettre en cause, des logiques comptables, administratives et bureaucratiques qui minent l'hôpital.

J'espère que la santé occupera une place centrale dans la campagne présidentielle. Les perceptions sur les questions de santé ont changé à l'issue de la crise : chacun a pu prendre la mesure de l'importance de ce service public, de ce bien qui a sauvé des vies et qui protège notre société. Nous espérons, avec l'appui de l'ensemble des professionnels du soin et du médico-social, réussir à tirer vers le haut les propositions qui seront faites à cette occasion, ce PLFSS ayant été un rendez-vous manqué. Pour ce faire, il convient de partir des besoins des territoires, de proposer d'entreprendre des réformes de fond, pour adapter ensuite nos arbitrages. À cet égard, À cet égard, nous avons largement répété que l'outil de régulation que constitue l'Ondam était dépassé. La maîtrise qu'il porte s'impose avant toute délibération sur les besoins en santé, dans nos territoires comme au Parlement.

ce PLFSS ne correspond toujours pas à ce que nous attendons d'une réelle politique de santé et de protection sociale. Le chemin qu'il nous faut prendre pour déterminer les besoins en santé de la Nation, pour mieux y répondre et endiguer définitivement cette crise profonde que vivent nos soignants, est celui de la démocratie. Le Parlement, les acteurs de santé, les élus locaux et nos concitoyens demandent à être associés à ces choix si fondamentaux pour notre collectivité nationale. Nous devons les entendre et agir en conséquence. En attendant de voir ce chemin se dessiner, nous voterons contre ce texte, dont nous considérons qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, des besoins et des réalités. Pendant deux ans, la sécurité sociale a maintenu et protégé notre société. Nous avons tous été personnellement témoins de son action concrète. Un consensus a été trouvé ici, dans nos rangs, sur l'aspect essentiel des métiers et des dispositifs qui nous ont permis de faire face. Tous ces discours doivent maintenant se traduire en actes pour mettre en oeuvre les réformes nécessaires et permettre à notre sécurité sociale d'assurer à l'avenir l'ensemble des missions de protection sociale dont notre démocratie peut être fière. La discussion

texte, la commission des affaires sociales, réunie ce matin, a décidé de proposer au Sénat d'opposer la question préalable sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En tout état de cause, nous prenons acte de la position de la majorité sénatoriale de s'exonérer d'un nouveau débat, et nous le regrettons. En effet, défendre le bicamérisme, c'est justement accepter le débat et les désaccords légitimes qui peuvent exister entre la majorité et l'opposition, ainsi qu'entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces désaccords ne sont pas nouveaux ; ils font partie du jeu démocratique et nous sommes capables de les surmonter, dans l'intérêt des Français. Défendre le bicamérisme, c'est aussi sortir des postures politiciennes, lorsqu'il s'agit de débattre du budget de la sécurité sociale, dont nous connaissons l'importance au quotidien pour nos concitoyens. Vous évoquez systématiquement la nécessité de respecter le Sénat, et nous partageons cette conviction. Mais pensez-vous que celui-ci sorte grandi de cette séquence budgétaire, lorsque les sénateurs s'exonèrent de leurs prérogatives et se privent de débattre sur les deux textes budgétaires en deux jours ? Vous défendez le bicamérisme dans toutes vos expressions publiques, mais dans les faits, vous le fragilisez par vos postures. Je sais que nous connaissons une séquence politique particulière ; le calendrier électoral intéresse d'ailleurs bien davantage les appareils politiques que les Français ... L'examen du budget ... L'examen du budget de la sécurité sociale, mes chers collègues, n'est ni le congrès des Républicains ni un énième lancement de campagne présidentielle avorté ! Soyons à la hauteur des enjeux et des défis qui attendent notre pays et auxquels le budget de la sécurité sociale apporte des réponses concrètes.

déplorent « l'absence de stratégie de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale à l'issue de la crise ». Mes chers collègues, vous êtes aveugles et sourds à ce qui se passe dans vos départements L'hôpital est au bord du gouffre, voire pire. Le plan blanc est utilisé pour rappeler le personnel et assurer l'activité quotidienne, alors qu'il est conçu pour faire face aux catastrophes naturelles ou aux attentats.

alors nous continuons à travailler. » Il n'est pas possible de continuer à rogner sur les dépenses de santé ! Il faut de nouvelles recettes pour la sécurité sociale, comme nous l'avons proposé. Or le Gouvernement

notre collègue Michelle Meunier a fait voter dans cet hémicycle un amendement visant à garantir aux personnes en situation de handicap le libre choix de leur fauteuil roulant.

proposition qui sera nécessaire dans l'avenir, au vu de la diminution du nombre de cotisants et de l'augmentation du nombre de retraités. La suppression par le Sénat de la trajectoire pluriannuelle des comptes sociaux est plus problématique, étant donné la persistance de la pandémie. Il faut revenir le plus vite possible à l'équilibre, sans sacrifier le financement de la santé, mais aussi sans augmenter les cotisations des entreprises afin de maintenir leur compétitivité et de favoriser l'emploi

pour financer leurs équipements, ce qui peut relever de la compétence de la sécurité sociale. Le Gouvernement renonce au plan Grand âge, sauf pour le maintien à domicile. C'est un début. Mais le texte ne prévoit pas une prise en charge suffisante de la dépendance en Ehpad pour les années

un beau débat sur le présent PLFSS. Il n'y avait pas de jeux de dupes, chacun défendait ses convictions et le ministre qui siégeait au banc expliquait la politique du Gouvernement. En revanche, monsieur Iacovelli,